séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. Nous reprenons la discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

voisins. En tant que sénateur du département de la Moselle, je serais favorable à une telle mesure, si elle correspondait à une logique administrative territoriale cohérente. Deux éléments ne me conviennent pas dans le système actuel. Premièrement, pour aménager l'autoroute A31

Mes chers collègues, si nous réussissons à donner aux Alsaciens ce département avec quelques compétences nouvelles qui seront peut-être utiles pour d'autres départements frontaliers, nous aurons réussi. Ayons donc ce débat sur la décentralisation au lieu de nous battre sur un nom qui va tromper les Alsaciens ; je pense qu'il faut leur dire la vérité. Ce que nous avons réussi est un pas, un petit pas. Mais le grand pas que nous devons à tous les Français, c'est une vraie décentralisation ; celle-là, nous ne l'avons pas

Venons-en à cette Arlésienne de l'écotaxe, à ce feuilleton parlementaire fait d'hésitations, voire d'errances gouvernementales, et qui n'est malheureusement pas clos. La demande alsacienne est plus que légitime. Nos voisins allemands ont mis en place une écotaxe en 2005. Depuis lors, le côté français du Rhin s'est trouvé saturé d'une noria de camions privilégiant un axe voisin gratuit. Je tiens à saluer très sérieusement la persévérance des collègues parlementaires qui, depuis seize ans, se battent pour parvenir enfin à un résultat tangible. Je les félicite d'autant plus que, depuis quatre ans que je suis sénateur, c'est le huitième texte de loi dans lequel je propose un dispositif similaire pour la Lorraine,

Oui, cette écotaxe alsacienne est nécessaire et légitime. Je salue MM. les rapporteurs Jean-Claude Anglars et Stéphane Le Rudulier,

l'examen du texte en commission, notre groupe a mis en garde contre le risque de faire payer le conducteur lorsque le propriétaire du véhicule fait défaut. Il n'y a aucune raison

sur l'axe Paris-Strasbourg, vous avez le choix entre l'autoroute A4, payante, et, quelques dizaines de kilomètres au sud, la nationale 4, gratuite. Résultat : 17 % de poids lourds

Je salue mes collègues Guillotin, Mizzon et Belrhiti, qui, dans une démarche transpartisane, nous ont rejoints au service de l'intérêt général. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre

validée à l'Assemblée nationale, puis que cette loi soit promulguée, puis qu'elle soit appliquée, puis que la région Grand Est s'attribue effectivement la compétence et, enfin, qu'elle l'applique.

de mettre en place l'écotaxe lorraine dès maintenant au profit de l'État serait de faciliter la décision d'enclencher les travaux de modernisation de cet axe saturé. En conclusion,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à mon tour à saluer les maires qui nous regardent, mais aussi les maires du département du Haut-Rhin qui sont présents dans les tribunes. à peine plus de deux ans, je m'exprimais ici même pour défendre et soutenir le souhait des Alsaciens et de leurs élus de donner une traduction institutionnelle à leur désir d'Alsace. L'Alsace souhaitait écrire une nouvelle page de son histoire, dans laquelle elle serait en capacité de mettre pleinement à profit ses spécificités, qu'elles soient linguistiques, géographiques ou encore culturelles. Aujourd'hui, au travers de la ratification de ces trois ordonnances, il nous est proposé de poursuivre un peu plus l'écriture de cette histoire. Il s'agit notamment de valider le cadre dans lequel la Collectivité européenne d'Alsace sera en mesure de mettre en place une redevance poids lourds. En conformité avec l'esprit de différenciation cher au Président de la République, la CEA pourra alors appréhender un peu plus son caractère frontalier et en tirer les conséquences.

Moi-même élue de ce territoire bordé par les trois frontières, je suis témoin des kilomètres de bouchons qui s'accumulent tous les jours sur l'A35 à la frontière suisse, en raison des camions qui cherchent à ne pas s'acquitter de la taxe allemande. S'agissant essentiellement de véhicules en transit, ce report de flux, non seulement ne génère aucune retombée économique positive pour le territoire, mais contribue largement à l'engorgement du trafic, est source de pollution atmosphérique et sonore, met en péril la sécurité des automobilistes et accélère l'usure des infrastructures. Il était donc plus que temps d'agir L'idée d'une telle taxe n'est pourtant pas nouvelle, puisque déjà en 2005 un amendement du député Yves Bur en prévoyait la mise en oeuvre à titre expérimental. Alors que cette taxe fut finalement abandonnée en 2013, en même temps que le projet national d'écotaxe, la CEA, grâce à l'important travail de coconstruction mené par ses élus avec le Gouvernement, sera prochainement en mesure, quant à elle, de faire aboutir ce projet. Alors que l'on parlait de disparition de l'Alsace, je veux dire ma fierté de voir celle-ci faire figure de précurseur

saisis, fruits d'un processus échappant largement aux logiques partisanes, traduisent les aspirations d'un territoire et de ses habitants. Aussi, le groupe RDPI s'exprimera en faveur de leur ratification. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais d'entrée me féliciter que nous soyons saisis d'un projet de loi de ratification des ordonnances prises sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 août 2019.

que les ordonnances prévues par cet article 13 soient prises un jour et qu'elles soient ratifiées. Une taxe touchant les poids lourds en transit avait déjà été votée pour l'Alsace par le Parlement contre l'avis du Gouvernement, mais celle-ci n'était jamais entrée en application faute des décrets d'application nécessaires. Chat échaudé craint l'eau froide, dit-on

Cet amendement avait recueilli l'assentiment de la commission des lois et il avait été voté par le Sénat, mais il fut ensuite rejeté à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, que faut-il penser des ordonnances que l'on nous propose de ratifier ? Ce sont bien entendu des textes techniques, et la première interrogation à cet égard est de savoir ce qu'en pensent celles et ceux qui auraient à les mettre en oeuvre, à savoir les élus de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est bien sûr ce qu'ont fait les rapporteurs des commissions concernées par le texte et les sénateurs alsaciens, dont je suis. Globalement, on peut dire que les textes qui nous sont soumis vont dans la bonne direction, monsieur le ministre. Des demandes complémentaires formulées par la Collectivité européenne d'Alsace ont été prises en compte par les rapporteurs et adoptées par les commissions concernées. Certes,

Oui, que cette taxe poids lourds soit mise en oeuvre au plus vite, c'est cette exigence, mes chers collègues, qui doit guider aujourd'hui le Sénat dans son appréhension du texte. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues lorrains, en particulier mosellans, il me semble qu'il ne faut pas profiter de ce projet de loi pour ouvrir, d'une façon ou d'une autre, le débat sur l'extension de la taxe à d'autres territoires, notamment au sillon lorrain.

qui a entraîné le transfert de tout le trafic poids lourds international de l'A5 allemande vers l'A35 en Alsace. Nous, sénateurs alsaciens, comme tous les Alsaciens, sommes aptes à en juger.

de retarder encore la mise en oeuvre du dispositif nécessaire à la résolution de ce problème est dangereux. Et si je puis me permettre, mes chers amis lorrains,

mes chers collègues, que penser de l'article 1 , introduit sur l'initiative des rapporteurs, qui prévoit une concertation avec les collectivités territoriales limitrophes en amont de la création de cette taxe ?

et sous la réserve explicite que cette concertation ne retarde pas la mise en oeuvre de la taxe, pourquoi s'y opposer ? Je terminerai en remerciant

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après en avoir été les demandeurs, puis les acteurs, allons-nous enfin, ce soir, être les spectateurs d'un retour à un fonctionnement normal de l'infrastructure routière que constitue l'A35 ? C'est en tout cas ce que nous, élus alsaciens, appelons de nos voeux. Voter en faveur de l'ordonnance qui instaure une contribution spécifique pour les transporteurs routiers permettra de répondre à une demande forte de la part de nombreux élus du territoire, que je salue, d'usagers et de riverains. Maire de Rixheim jusqu'en 2020, je connais parfaitement le sujet, puisque cette autoroute est tangente à ma commune, et il n'est pas exagéré de dire que la situation est devenue insupportable et dangereuse, avec des ralentissements, des bouchons et de nombreux accidents en tout genre.

gouvernement Schröder, les transporteurs préfèrent éviter l'autoroute A5 allemande : ils choisissent de modifier leur trajet et de bifurquer vers l'autoroute alsacienne située à seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau. C'est l'effet de bord de cette taxe instituée outre-Rhin qui a contribué à la saturation de notre réseau autoroutier. Depuis plus de quinze ans, nous, élus locaux, souhaitons l'instauration d'une redevance poids lourds pour lutter contre cette inflation du trafic autoroutier. Depuis sa création, la Collectivité européenne d'Alsace a la capacité légale de mettre en place une taxe sur les poids lourds, l'ordonnance du 26 mai 2021 en fixant les modalités d'application et laissant une certaine latitude à l'exécutif local, avec une liberté de définir le réseau taxé, les tarifs ou encore l'organisation. L'idée générale des élus est bien de cibler le transport transfrontalier de marchandises qui passe par notre territoire sans y livrer véritablement de produits. Il faut absolument éviter trop de reports de l'Allemagne et de la Suisse vers la France. Cette taxe poids lourds ne doit pas être vécue comme une arme fiscale pénalisant nos transporteurs routiers ou les utilisateurs de camions côté alsacien. Elle doit permettre au contraire une meilleure répartition des flux de poids lourds.

Cette contribution permettra à terme de favoriser l'émergence d'une flotte de camions moins polluants, plus vertueux, et soutiendra l'émergence du fret ferroviaire et fluvial. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous favorables ici à l'instauration de cette taxe, fruit d'une étroite concertation entre la Collectivité européenne d'Alsace, le Gouvernement et les élus locaux. Vous le voyez, mes chers collègues, cette initiative, qui n'est pas une fin en soi, mais bien un projet pilote, comme l'a rappelé André Reichardt, est appelée à terme à être appliquée là où elle sera nécessaire, y compris en Lorraine. C'est une initiative qui va dans le bon sens. C'est un projet cohérent et pragmatique, qui doit résoudre la difficile équation de désengorger notre autoroute tout en prenant soin de ne pas pénaliser nos acteurs économiques locaux. Ce projet permet de travailler concrètement à la mise en place de solutions de rechange durables et responsables.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Collectivité européenne d'Alsace (CEA) a la compétence d'instaurer une taxe sur son domaine routier et autoroutier depuis le 1 janvier 2021, afin de contrer la taxe allemande qui a renvoyé les flux de camions vers l'Alsace et le sillon rhénan français. Cela règle un problème propre à la CEA, et je comprends et soutiens la réaction des Alsaciens face à ce problème. Toutefois, je ne vois pas comment le trafic des camions venant d'Allemagne se déporterait vers la Moselle, obligeant les transporteurs à effectuer un détour de plus de 150

Je tiens à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le danger que peut représenter cette taxe pour l'économie locale de la région Grand Est.

sur le seul territoire alsacien aura pour principale conséquence le déport d'une partie du trafic sur l'autoroute de Lorraine A31, déjà saturée par un flux continu de poids lourds et cause de multiples nuisances- pollution sonore, émissions de gaz à effet de serre, congestion routière, etc. C'est déjà la réalité Même si la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets permet au Gouvernement de légiférer par ordonnances, durant un délai de deux ans, pour permettre aux régions de mettre en place des contributions spécifiques sur le transport routier de marchandises, il faut agir sans attendre, pour que, dans l'intervalle, l'État puisse instaurer une taxe poids lourds sur l'autoroute A31. J'ai beaucoup de mal à comprendre que cette logique ne soit pas partagée par l'ensemble des sénateurs mosellans.

Ensuite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ... Il semble en effet important pour la région Grand Est, comme l'a fait la CEA, de prendre le temps d'élaborer son dispositif en coconstruction avec les services de l'État.

Un certain nombre de modalités relèvent du domaine de la loi : l'assiette, les taux et les modalités de recouvrement. S'agissant de l'amendement n° 4, sa rédaction laisse penser que la région Grand Est pourrait instituer une taxe sur des voies dont elle n'est pas propriétaire actuellement. Ces axes relèvent, pour l'heure du moins, de l'État ; il est donc prématuré de donner une suite favorable à cette proposition.

L'Alsace est une terre d'expérimentation. Elle fera donc le travail pour vous, en essuyant peut-être les plâtres, parce que la mise en place n'est pas aussi facile que cela. En même temps-

Jacquin. Je ne parlerai pas de la Lorraine. J'essaie d'apaiser les esprits ... C'est plus en connaisseur de la question des transports que je vous alerte, mes chers amis alsaciens, sur un risque particulier.

Les VUL, ce sont ces petits camions bâchés qui permettent aux transporteurs, bien souvent des pays de l'Est- c'est une réalité ! -, de s'affranchir des chronotachygraphes, des limitations de tonnage en ville

Quel est l'avis de la commission ? La question se pose d'intégrer de possibles évolutions relatives au champ des véhicules taxables, notamment au regard de l'extension du périmètre de la directive européenne à l'occasion de sa prochaine révision, qui pourrait concerner les véhicules utilitaires légers. Comme l'a indiqué M. Jacquin, la commission a souhaité anticiper la révision de la directive Eurovignette en introduisant un article 1 , qui permettra à la CEA, si la révision de la directive va dans ce sens, de prendre en compte des émissions de CO2 pour la définition du taux de la taxe qu'elle aura mise mise en place. Cette même logique pourrait donc nous conduire à anticiper d'autres éventuelles évolutions. Néanmoins, d'après les acteurs interrogés, le contournement de la taxe par le recours aux camionnettes est, du moins pour l'heure, un problème de second ordre. C'est pourquoi la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

vote. L'objet de cet amendement me paraît particulièrement pertinent. Je pense en effet que l'amplitude de la marge dans laquelle la CEA choisira le tonnage à partir duquel se déclenchera la taxe,

peuplée. Dans la mesure où les taxes pourraient se multiplier à l'avenir, il est nécessaire de sécuriser cette définition, sauf à créer des ruptures d'égalité entre les territoires, qui pourraient décider ce qui doit être considéré comme une zone peuplée. Enfin, cet article contraint l'État à définir la méthode d'évaluation des coûts engendrés par la pollution. Cela signifie non pas que la CEA devra mettre en place la majoration pour coûts externes, mais bien plutôt que l'État devra l'éclairer sur la méthode à suivre, si elle souhaite l'instituer. L'article 1 constitue donc un apport dont il serait dommage de se priver, d'autant qu'il vise à permettre à la CEA de mieux exercer ses responsabilités. En conséquence, la commission émet un avis défavorable

La commission a d'ores et déjà souhaité réduire les conditions dans lesquelles le conducteur peut être considéré comme solidairement responsable du paiement de la taxe, en prévoyant que cela ne peut arriver qu'en dernier ressort.

nous entendons vos réticences et les partageons : les conducteurs sont souvent des salariés d'entreprises de transport. Il ne leur revient pas d'assumer le paiement de la taxe. C'est pourquoi, sur cet amendement,

cela a été rappelé, il s'agit d'un dispositif à vocation subsidiaire, qui paraît nécessaire à la responsabilisation des redevables. Le Gouvernement est favorable au maintien du dispositif, celui-ci ayant déjà été modifié par la commission saisie

l'avis de la commission ? La commission a souhaité introduire une procédure de régularisation sans pénalité au bénéfice des seuls redevables occasionnels de la taxe. Cette mesure est un progrès pour trois raisons. Premièrement, il s'agit d'un dispositif inspiré du modèle allemand, dont les modalités sont encadrées. Ainsi, le redevable aurait deux jours pour régulariser sa situation et il ne devrait avoir fait l'objet d'aucune constatation d'infraction dans les six derniers mois. Deuxièmement, il s'agit de donner une certaine souplesse au dispositif de sanction, dans une logique de « droit à l'erreur ». Ainsi, les redevables occasionnels pourraient, en toute bonne foi, avoir oublié de s'acquitter de la taxe. Troisièmement, il s'agit d'une possibilité offerte à la CEA, qu'elle est libre d'utiliser ou non.

la commission est défavorable à la suppression de l'article 1, introduit sur l'initiative de la commission des lois, qui permet de faciliter le recouvrement des amendes prononcées ainsi que de la somme due au titre de la taxe, afin d'en garantir le rendement. Il s'agit d'ailleurs d'une possibilité offerte à la CEA, qu'elle est libre d'utiliser ou non. L'idée est de faire de cette ordonnance un modèle transposable dans l'avenir. Chaque collectivité pourra ainsi, sur cette base, choisir les modalités de mise en oeuvre qui lui correspondent le plus. La parole est à M. le

? La commission a cherché à préciser les dispositions relatives au contrôle automatique du respect des dispositions régissant la taxe, en se fondant sur le modèle existant pour les pour les ZFE, notamment en ouvrant aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu'aux agents assermentés de la CEA la possibilité de mettre en oeuvre ces dispositifs. Il s'agit encore une fois d'une possibilité offerte à la CEA, qu'elle est libre d'activer ou non.

de dépenser de la manière qu'elle jugera la plus pertinente. Je comprends le principe de cet amendement. Dans la mesure où il s'agit d'une taxe environnementale, il serait opportun que son produit serve à financer des dépenses vertueuses. Pour autant, fixer dans la loi les possibilités de dépenses de cette taxe par la CEA ne paraît pas opportun pour deux raisons. D'une part, la CEA est libre de dépenser ces montants comme elle le souhaite, sur le fondement de la libre administration des collectivités territoriales et de leur autonomie financière.

mais prévoir au plus six ans n'est ni justifié ni politiquement acceptable. Un délai de trois ans est suffisant : il s'inscrirait dans la perspective d'une entrée en vigueur vers 2023 ou 2024. L'échéance de 2024 serait d'ailleurs réaliste. Elle répondrait à la fois à la volonté largement consensuelle de la population et aux nécessités pragmatiques de la concertation et de la mise en oeuvre. Ce dossier alsacien souffre depuis seize ans de procrastination publique chronique : il est essentiel de signifier clairement par cette ordonnance la volonté nouvelle d'aboutir. Nous appelons donc à prendre en considération les attentes des habitants du territoire alsacien en fixant l'entrée en vigueur de la taxe à une date antérieure à trois ans à compter de la publication de l'ordonnance.

Pour autant, réduire de moitié le temps imparti à la CEA pourrait avoir un effet contre-productif, soit en la contraignant à instituer la taxe de manière précipitée, soit en l'empêchant tout simplement de la mettre en place si les délais de mise en oeuvre se révélaient plus longs que prévu. Il me semble que ce n'est pas l'effet que vous recherchez, De plus, le délai de six ans fixé par l'article 56 de l'ordonnance est un délai maximal. Si la CEA est prête avant cette échéance, je ne doute pas qu'elle mettra en place cette taxe avant la fin du délai imparti. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Quel est l'avis de la commission ? Les chargeurs jouent en effet un rôle fondamental dans la définition des schémas de transport. Il semble donc bienvenu de les consulter en amont de la mise en place de la taxe, au même titre que les transporteurs. De plus, la CEA nous a indiqué qu'elle comptait d'ores et déjà les consulter. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

l'État pourrait considérer qu'une telle taxe n'est en réalité pas nécessaire, les reports de trafics pouvant être négligeables. L'article 61 de l'ordonnance prévoit que le Gouvernement remette au Parlement un rapport au plus tard cinq ans après la mise en oeuvre de la taxe présentant le bilan de la taxe sur la maîtrise du trafic routier de marchandises sur le territoire de la CEA. Sur l'initiative de son rapporteur, la commission du développement durable a judicieusement complété le contenu de ce rapport : celui-ci devra évaluer les éventuels reports de trafic que pourrait entraîner la mise en oeuvre d'une taxe sur le transport de marchandises. Elle a également prévu tout aussi judicieusement d'y ajouter un rapport d'étape au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la taxe. Cet amendement vise à préciser que ce rapport d'étape doit comprendre une évaluation des reports de trafic sur sur l'A31, laquelle permettra au Gouvernement de disposer des éléments nécessaires pour juger de l'opportunité ou non de mettre en oeuvre une taxe sur cet

évalue les reports de trafic sur le réseau du domaine public des régions, des départements et des communes limitrophes. Les reports sur l'A31 seront donc bien évalués. Par conséquent, la

amendement. Je souhaite donc que, en signe de solidarité, nos amis alsaciens, nombreux ce soir, votent cette disposition.

que nous n'aimerions pas que les principes qui ont été retenus ici nous soient appliqués- fort heureusement, personne ne l'a réclamé. L'enseignement que j'en tire, c'est la confirmation

prises sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public

Le Sénat a adopté.